Pour pallier les difficultés qu'il a lui-même créées des politiques antisociales, comme la baisse des aides personnalisées au logement (APL) ou la réforme de l'assurance chômage, le Gouvernement multiplie les primes désocialisées et défiscalisées, qui grèvent les comptes publics, encourageant de fait les entreprises à substituer le salaire variable aux augmentations générales pérennes. À l'opposé, de nombreux pays augmentent le salaire horaire minimum. Ainsi, l'Allemagne le portera à 12 euros

vivre dignement et satisfaire ses besoins essentiels, les écologistes soutiennent l'augmentation du SMIC, car il n'est pas tolérable que la figure du travailleur pauvre s'étende dans notre pays. La parole

vous voulez augmenter le pouvoir d'achat des Françaises et des Français ? Vous voulez rétablir la valeur travail ? Vous voulez en finir avec les filières qui n'arrivent pas à recruter ? Nous avons la solution : porter le SMIC à 1 500 euros

nous faisons davantage contribuer les entreprises. En 2021, notre pays comptait 2 millions de salariés rémunérés au SMIC, soit 12 % des salariés du secteur privé, parmi lesquels une grande majorité de femmes.

dans la continuité des politiques menées à l'étranger pour améliorer le pouvoir d'achat. Le salaire minimum a connu une augmentation de plus de 30 % en Espagne et de plus de 25 % en Allemagne. Au Royaume-Uni, il est désormais plus haut que le SMIC.

aux premiers de corvée- je devrais plutôt dire aux premières de corvée -, alors que les entreprises du CAC 40, aux profits record de 160 milliards d'euros en 2020, ne sont pas mises à contribution ! La parole

qui défend les intérêts des travailleuses et des travailleurs et d'un gouvernement et d'une droite qui se retrouvent pour refuser l'augmentation du SMIC.

monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour examiner le fameux article 1 de ce projet de loi, qui est la traduction législative de la fameuse prime dite Macron.

Sous couvert d'une augmentation du pouvoir d'achat d'une partie des Français, vous mettez en place une incitation à ne pas augmenter les salaires, et vous accélérez la fragilisation, déjà bien entamée sous le précédent quinquennat, de notre système de protection sociale. Je m'explique : un employeur qui a le choix entre augmenter les salaires ou verser une prime défiscalisée et sans cotisations sociales choisira la solution la moins coûteuse et la moins pérenne. Vous créez donc un effet d'aubaine qui ne bénéficiera pas aux salariés. aux salariés. En outre, avec un tel dispositif, vous dites une chose : le travail coûte trop cher, car la protection sociale des Français coûte trop cher. La défiscalisation et la désocialisation des primes n'auront qu'un effet limité, sur un temps très court, pour les Français. En revanche, l'effet à long terme sur les finances publiques est bien réel. Quand on supprime les cotisations sociales et que l'on défiscalise, on prive de recettes la protection sociale et le budget de l'État. Venant d'un gouvernement qui veut renflouer les caisses en réduisant les droits des chômeurs et en augmentant de trois ans la durée de cotisation ouvrant des droits à la retraite, c'est indigne, monsieur le ministre ! Vous organisez donc la casse du système pour constater à terme qu'il ne marche plus. Vous êtes, de fait, les fossoyeurs des jours heureux du Conseil national de la Résistance. Encore une fois, je vous demande d'organiser une conférence salariale à la rentrée. Chaque Français doit vivre dignement du fruit de son travail. Tout le reste n'est que tromperie cynique.

On ne vit pas avec un SMIC ; on survit. Avec l'explosion de l'inflation, on survit encore plus difficilement. Il est donc urgent de mettre en place des mesures pour contenir les effets de l'augmentation des prix sur les classes moyennes et les plus précaires. Or le présent projet de loi ne permet ne prévoit que des dispositions de court terme, aux effets incertains. Ainsi, selon l'étude d'impact réalisée par l'Assemblée nationale, il est « probable » qu'un plus grand nombre de salariés seront concernés par cette prime. Or je rappelle que seuls 6 millions de salariés, sur un total de 25 millions, ont bénéficié des anciennes versions de la prime, pour des montants très éloignés des plafonds autorisés. Combien de nouveaux salariés pourront prétendre à cette nouvelle prime ? Trop peu ! C'est une certitude. La solution à la crise inflationniste n'est pas dans ce texte. Seule une véritable politique de revalorisation des salaires permettrait à de nombreux Français de vivre de leur travail dignement. Je suis également décontenancée par l'exonération de cotisations sur cette prime pour les groupes ayant réalisé des profits records lors de l'épidémie de la covid-19 ou ayant des filiales installées dans des paradis fiscaux,

politiques. Vous refusez ainsi que les salariés puissent gagner au minimum 1 500 euros. Pour le Gouvernement et pour les droites, le partage de la valeur consiste en deux choses : inciter les employeurs à verser des primes et faciliter la mise en place de l'intéressement en entreprise. Pour les salariés qui n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois, le versement d'une prime peut sembler être une bonne nouvelle. Mais si une prime

exonérations, ce sont près de 600 millions d'euros en moins pour nos services publics, nos écoles. Nous disons donc : « Attention à l'effet boomerang ! » Avec ces dispositifs, le Gouvernement a réussi à se mettre à dos ses propres supporters. Dans une tribune publiée le 23 juillet dans, l'Institut Montaigne a ainsi critiqué vos primes et appelé à revaloriser l'intéressement et la participation en entreprise. Heureusement, les droites sénatoriales sont intervenues en commission contre la cannibalisation de l'intéressement et la participation ». La prime Macron a bénéficié à 5 millions de salariés entre 2021 et 2022, pour un montant moyen de 545 euros. Ce n'est pas la peine de donner l'illusion aux salariés qu'ils auront 6 000 euros de primes. C'est une vaste blague

Ces derniers mois, les conflits sociaux se sont partout multipliés afin d'obtenir des revalorisations salariales au moins à la hauteur du taux d'inflation, qui sera encore plus élevé à la rentrée, et vous le savez

Face à l'urgence, une succession de mesures ponctuelles et majoritairement financées par l'État ne peut en aucun cas constituer une réponse suffisante. On ne trouve nulle part trace de partage de la richesse ni même du fameux « ruissellement Le CAC 40 ayant dégagé près de 160 milliards d'euros de bénéfices en 2021 et versé près de 60 milliards d'euros de dividendes, il est fort regrettable que la question de l'augmentation des salaires soit constamment éludée. Comment justifier que les salariés, en particulier ceux au SMIC ou juste au-dessus, s'appauvrissent d'année en année ? Comment justifier que le Gouvernement refuse d'appeler à la solidarité nationale de tous, y compris de celles et ceux qui se sont le plus enrichis au cours des derniers mois ? Mme la Première ministre Élisabeth Borne nous avait indiqué que les organisations syndicales et patronales trouveraient en elle une interlocutrice « franche, constructive et déterminée ». Mais que demandent tous les syndicats aujourd'hui ? L'ouverture de discussions sur les salaires ! Et quel compromis bâtit le Gouvernement avec eux ? Aucun La prise en charge de mesures en faveur du pouvoir d'achat relève aussi de la responsabilité des employeurs. Elle doit se traduire par une augmentation des salaires. Il serait grand temps que ce gouvernement l'entende

Or la crise sanitaire a provoqué une crise économique dont les effets dévastateurs sont durables et se font toujours sentir. Certains secteurs, comme celui du tourisme, dans lequel exercent nombre de nos compatriotes à l'étranger, mais également les artisans et les petits entrepreneurs continuent de subir le contrecoup des confinements et de la fermeture des frontières. Alors que les entreprises implantées sur le territoire national ont bénéficié d'un soutien exceptionnel, celles qui sont implantées à l'étranger n'ont pas été intégrées dans le périmètre du plan de relance. Tous les acteurs économiques l'ont regretté. Nous l'avons d'ailleurs déjà dit dans cet hémicycle en adoptant l'année dernière au Sénat, une proposition de loi présentée par notre ancienne collègue Jacky Deromedi. Les conseillers du commerce extérieur, ainsi que le réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'étranger ont également créé une structure, EFE International, afin de soutenir les entreprises françaises à l'étranger qui travaillent la marque France. Cette structure mériterait tout notre soutien. Par ailleurs, le secours occasionnel de solidarité mis en place par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères au mois d'avril 2020 en faveur de nos compatriotes ayant subi une diminution substantielle de leurs revenus à cause de la pandémie prendra fin le 31 août prochain. À cela s'ajoute la flambée des prix, notamment de l'énergie et des denrées alimentaires, qui n'épargne aucun continent. Si ce projet de loi prévoit une revalorisation de 4 % des prestations sociales et des pensions de retraite, rien n'est prévu pour nos compatriotes établis hors de France.

Cozic, sur l'article. Monsieur le ministre, ces cinq dernières années, le Gouvernement a considéré que la lutte contre la pauvreté passait avant tout par le renforcement des incitations à travailler. Sur le fond, je ne peux qu'acquiescer. En revanche, sur la forme, nos chemins divergent. Car, pour y parvenir, vous misez systématiquement sur des dispositifs qui ne touchent pas aux salaires ; ce n'est pas nouveau. Vous avez ainsi incité les entreprises à verser des primes exceptionnelles en 2018, en 2020 ou à développer la part variable des salaires

telle stratégie n'est pas viable sur le temps long terme. Elle crée des effets d'aubaine pour les entreprises. En effet, à court terme, leurs salariés touchent plus pour un coût maîtrisé, mais à long terme, les salaires restent bas. Les salariés sont, eux, perdants sur presque tous les plans. Leurs revenus deviennent imprévisibles. D'abord, une aide distribuée par l'État peut disparaître à tout moment, alors qu'un salaire ne peut être baissé de façon unilatérale par l'employeur. Ensuite, leur progression salariale de carrière est nécessairement ralentie. Enfin, ils cotisent moins pour leur retraite, car ces revenus ne sont pas soumis à cotisations sociales. Monsieur le ministre, acceptez un débat clair et juste sur le sujet. SER vous propose de convoquer un Grenelle des salaires réunissant à la rentrée les partenaires sociaux et patronaux, l'État et les parlementaires pour discuter de la juste répartition des salaires et, incidemment, de l'augmentation des plus bas d'entre eux.

et d'une part brute. Les cotisations patronales sont des salaires différés, qui permettent de financer notre modèle social et la sécurité sociale, auxquels d'ailleurs vous voulez vous attaquer avec votre projet de grande sécurité sociale, qui n'a rien à voir avec la prime d'activité. Vous donnez de la main gauche et vous reprenez de la main droite avec l'impôt

et, à terme, de la protection sociale de tous les Français. Les cotisations sociales sont des salaires différés ; je l'ai dit précédemment. C'est pourquoi nous vous proposons de taxer les grands groupes profiteurs de crise pour financer les primes Macron aléatoires et discrétionnaires ou, à défaut, de resocialiser ces primes, qui ne bénéficient qu'à quelques-uns, afin qu'elles ne soient pas financées par la baisse des droits sociaux de tous.

Actuellement, la PPV peut être versée en plusieurs tranches, mais elle ne peut être décidée qu'une fois l'an. Si, d'ordinaire, la majorité des entreprises ont peu de visibilité sur la réalisation de leur chiffre d'affaires et sur leur situation financière en cours d'année, dans la conjoncture économique incertaine que nous connaissons, la prévision devient ardue. Elles sont donc contraintes soit de limiter le montant de la PPV à un montant le moins risqué possible, soit d'attendre la fin de la période d'attribution pour s'assurer de leur capacité à la verser. Le mécanisme de la PPV pourrait être adapté pour permettre à l'employeur de verser une ou plusieurs PPV durant la période de référence, dans la limite du montant du plafond global de la PPV déjà fixé par la loi, en veillant à ne pas procéder à des versements mensuels assimilables

à l'employeur de verser une ou plusieurs primes durant la période de référence, dans la limite du plafond global fixé par le projet de loi. Cette adaptation permettrait aux salariés de bénéficier de primes plus élevées sans attendre la fin de la période.

pour les entreprises de moins de cinquante salariés. Le Gouvernement souhaite que ce dispositif nouveau de partage de la valeur puisse concerner toutes les entreprises, et ce au-delà du 31 décembre 2023. L'amendement n° 22, présenté

au service de l'intérêt général. Ce secteur constitue la réponse aux besoins de vie du quotidien et organise l'emploi de proximité qualifié et solidaire. Or une ambiguïté subsiste quant à l'éligibilité des millions de salariés de particuliers employeurs à la PPV instituée par l'article 1 du projet de loi. L'emploi direct à domicile représentant une masse salariale

dont 0,3 point de pur effet d'aubaine. Sans une telle mesure, la part concernée aurait donné lieu à cotisations, impôts, droits contributifs et augmentation pérenne du salaire. L'Insee constate également que les salaires « progressent moins vite dans les entreprises ayant versé une prime que dans celles qui s'en abstiennent

Le Conseil d'État ne s'y est pas trompé : « [ ...] la liberté de choix laissée à l'employeur dans la répartition de la " prime de partage de la valeur " [ ...] ne permet pas de garantir qu'elle contribuera effectivement à la protection du pouvoir d'achat et, en particulier, qu'elle bénéficiera substantiellement aux plus bas salaires. du Conseil d'État, et non simplement de la gauche de l'hémicycle ... Or la lutte contre l'insécurité sociale résultant d'une inflation galopante devrait renforcer plutôt la résilience collective. Après tant d'alertes, cet amendement a pour objet de conditionner l'exonération de la PPV à la conclusion d'un accord d'entreprise portant sur la revalorisation de l'ensemble

que nous connaissons. Si nous pensons fort justement aux salariés, aux ouvriers, à toutes celles et tous ceux qui ont des contrats dits classiques et qui entrent dans les critères de conditionnalité, il m'apparaît pourtant nécessaire- le constat est partagé par l'ensemble des signataires de cet amendement -de ne pas oublier certains travailleurs,

code de l'éducation. La prime n'est pas une obligation pour l'employeur, mais la désocialisation et la défiscalisation sont particulièrement incitatives. Je tiens à ce qu'elles le soient pour le plus grand nombre, afin de donner à l'employeur la possibilité de donner un coup de pouce au-delà du minimum légal qui est la plupart du temps prévu dans ces contrats. C'est une manière de récompenser les efforts déployés. Nous devons y veiller, car c'est une question de justice sociale et un devoir commun que de soutenir nos jeunes, notre avenir.

Les revalorisations salariales, tous dispositifs confondus, s'élèvent, selon les secteurs et les tailles d'entreprise, de 5 % à 10 % en 2022. Afin d'encourager cette mobilisation, notre amendement vise à leur permettre de verser une prime universelle exceptionnelle défiscalisée et désocialisée, allant jusqu'à 2 000 euros, à l'ensemble de leurs salariés, quel que soit leur niveau de rémunération. L'exonération du forfait social serait ainsi maintenue pour une première tranche de distribution allant jusqu'à 2 000 euros. Au-delà, le régime fiscal et social du dispositif pérenne de prime de pouvoir d'achat s'appliquerait. Alors que deux tiers des ETI envisagent de verser une prime de pouvoir d'achat en 2022 et ont à coeur de préserver la cohésion du collectif en traitant équitablement l'ensemble de leurs salariés, la coexistence de deux régimes de primes suivant le niveau de rémunération et, singulièrement, l'assujettissement au forfait social d'une partie des primes, sont de nature à brider le recours à ce dispositif exceptionnel et à amputer les montants distribués.

Cet amendement vise donc à mettre en oeuvre une prime universelle, défiscalisée et désocialisée, d'un montant maximum de 2 000 euros, à destination de l'ensemble des salariés des PME et des ETI, pour répondre aux problématiques de pouvoir d'achat dans un contexte économique inflationniste. Cet amendement tend, d'une part, à permettre aux employeurs d'attribuer une prime défiscalisée de façon trimestrielle plutôt qu'annuelle et, d'autre part, à doubler son montant pour l'année. Cela permettra aux salariés d'avoir un budget plus en adéquation avec leurs besoins.

-pour que les compensations soient totalement financées par l'État, conformément d'ailleurs au code de la sécurité sociale. Mais, dès lors que vous exonérez de cotisations sociales, c'est un manque à gagner. Vous le comblez avec de l'argent de l'État

particulière soit portée à l'égalité salariale. Mais j'ai l'impression que ce gouvernement, finalement, ressemble trait pour trait au précédent et que, malgré les belles promesses de changement, les femmes vont devoir encore attendre, souffrir et lutter. lutter. Franchement, face à l'urgence et à la gravité de la situation, notre amendement est plutôt modéré, puisqu'il tend uniquement à instaurer comme condition au maintien des exonérations sociales de la PPV l'ouverture de négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tous les ans. C'est tout de même la moindre des choses. J'espère

des entreprises ayant un recours abusif aux contrats à temps partiel. Il y a un risque d'effet d'aubaine, alors que les employés à temps partiel sont déjà frappés d'une double peine

Cette précarité subie est particulièrement fréquente chez les femmes, titulaires de 80 % des emplois à temps partiel. Il est indispensable d'encourager les entreprises à recruter à temps complet et d'éviter de soutenir indirectement les entreprises qui recrutent majoritairement à temps partiel. C'est pourquoi notre amendement vise à exclure du bénéfice des exonérations de cotisations sociales les entreprises où les contrats à temps partiel représentent plus de 20 % de la masse salariale totale.

Son montant peut aller jusqu'à 3 000 euros par bénéficiaire et par année, et jusqu'à 6 000 euros lorsque la PPV est versée par une entreprise qui met en oeuvre un dispositif d'intéressement, par un organisme d'intérêt général ou, s'agissant des primes versées aux travailleurs handicapés, par un établissement ou un service d'aide par le travail. De fait, de tels dispositifs restent compliqués à mettre en oeuvre pour les entreprises de proximité, dont l'immense majorité comptent moins de cinquante salariés, notamment parce qu'ils engagent l'entreprise sur trois ans, dans un contexte où les bénéfices d'une année n ne sauraient être garantis pour l'année ni,, ni,, pour l'année . Cet amendement s'inspire de l'esprit de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021, qui autorise les entreprises de moins de cinquante salariés à verser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat jusqu'à un montant de 2 000 euros, sans condition liée à la mise en oeuvre d'un dispositif d'intéressement, au même titre que les associations et les fondations mentionnées aux a) et b) du 1° des articles 200 et 238 du code général des impôts. L'amendement : La parole est à M. Olivier Henno. Cet amendement vise à supprimer pour les TPE la condition de mise en place d'un dispositif d'intéressement pour accéder à un montant de prime revalorisé à 6 000 euros. En effet, l'obligation de conclure un accord d'intéressement peut représenter une contrainte administrative dissuasive pour ces très petites entreprises de moins de dix salariés,

Les accords d'intéressement sont un outil qui lie les salariés à la performance et, souvent, à la rentabilité de l'entreprise. Mais la hausse des bénéfices de l'entreprise doit permettre une augmentation des salaires, de la même manière qu'elle aboutit actuellement à une augmentation spectaculaire et continue de la rémunération des P-DG. En 2021, selon

Selon l'Insee, au mois de décembre 2021, le taux de marge des entreprises s'est envolé aux alentours de 36 %, son plus haut niveau depuis 1949. Cette augmentation n'est pas le fruit du hasard. Elle a été permise par la décorrélation, dans les années 1980, entre les salaires et l'inflation, diminution de la part des salaires dans le PIB, tandis que les taux de marge des entreprises ne cessent, eux, d'atteindre des records chaque année. Car il s'agit bien du partage des richesses créées. La compression de la part de rémunération du travail

les dispositifs existants d'épargne salariale. Un tel effet de bord contreviendrait à la volonté affichée par le Gouvernement de promouvoir et développer ceux-ci, au premier rang desquels l'intéressement. En effet, la PEPA, comme les dispositifs d'épargne salariale, n'a vocation à se substituer à aucun élément de rémunération. L'épargne salariale demeure essentiellement financée par les flux versés par l'entreprise : participation, intéressement, abondement. Ses frais sont pris en charge par l'entreprise et elle constitue pour de nombreux salariés leur seule épargne financière. C'est une épargne majoritairement investie en actions et obligations privées, qui finance les entreprises. Cette tendance a été accentuée par la loi Pacte, qui a fléché une part des investissements vers les fonds dits PEA-PME. En instaurant la PEPA, dont les caractéristiques font référence au cadre légal de l'épargne salariale, le Gouvernement introduit une concurrence avec la prime d'intéressement et prend le risque d'une éviction de l'intéressement au profit de cette nouvelle prime, ce qui pénalisera le financement de l'économie productive. La PEPA favorise le court terme et la consommation de biens importés, alors que les dispositifs d'épargne salariale permettent le financement à long terme de nos entreprises. C'est pourquoi cet amendement vise à exonérer d'impôts et de cotisations sociales tous les versements de la PEPA sur les dispositifs d'épargne salariale, et ce sans condition de rémunération.

D'abord, nous traitons d'une prime de partage de la valeur : dès lors que l'amendement concerne les particuliers employeurs dans une relation avec des salariés à domicile, cette notion de partage de la valeur perd un peu de sens. Ensuite, nous reconduisons

n° 90 rectifié proposent d'appliquer les taux de l'entreprise utilisatrice plutôt que ceux de l'entreprise de travail temporaire. Or l'intégralité des exonérations de cotisations- calcul de crédit d'impôt, dispositif d'intervention de l'État,

les modalités de calcul de l'intégralité des dispositions, non plus en fonction de l'entreprise de travail temporaire, mais en fonction de l'entreprise utilisatrice. Avis défavorable. Avis défavorable sur les amendements n 151, 152 et 153, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure,

coordination, monsieur le président.

de loi. Si l'intention du Gouvernement d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés est louable, sa proposition crée un manque à gagner pour les organismes de sécurité sociale tant il est prouvé que ces dispositifs de prime et d'intéressement se substituent, de fait, dans un certain nombre d'entreprises, à la rémunération de base. Or le Gouvernement ne propose pas de compenser ce manque à gagner, alors que la sécurité sociale a enregistré, en 2021, un déficit de 31,2 milliards d'euros.

Cet amendement tend à ajouter un critère de performance individuelle aux quatre critères déjà prévus dans le projet de loi afin d'attribuer la prime de partage de la valeur de manière justifiée

de bénéficier de plus de flexibilité quant au versement de la prime de partage de la valeur. Le mode de fonctionnement des TPE est loin de celui des PME ou des grandes entreprises. Du fait du très petit nombre de salariés concernés, il semble opportun que le chef d'entreprise puisse individualiser le versement de la prime. À ce titre, en intégrant le critère de performance individuelle aux quatre autres prévus par le texte, cette prime pourrait récompenser un ou plusieurs

Ils ont rejeté du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail, comme l'a souligné Philippe Mouiller. Ces critères de modulation sont importants, puisqu'ils permettent d'adapter le dispositif de manière suffisamment fine en fonction de la situation du bénéficiaire et de son implication au sein de l'entreprise. Comme vous le savez, j'ai soutenu l'ouverture de cette prime à d'autres types de contrats. Je pense que nous devons aller plus loin sur la question des personnes en situation d'insertion afin de valoriser

Poncet Monge. Cet amendement, déposé par ma collègue Mélanie Vogel, vise à lutter contre les inégalités de genre au sein de l'entreprise. Les femmes sont souvent dans une situation économique précaire, alors même que les métiers précarisés où elles sont majoritaires sont essentiels à notre société. Ces dynamiques sont bien documentées par les sciences humaines. L'assignation des femmes à la sphère domestique et au travail non rémunéré participe largement du fait que, historiquement, les réseaux de pouvoir sont quasi exclusivement masculins

En l'absence de disposition spécifique, la prime mentionnée à l'article 1 ne remédiera pas aux inégalités de genres Ainsi, selon l'Insee, les femmes occupent 79 % des emplois à temps partiel- souvent subis -, 70 % des emplois à bas salaires et 59 % des emplois payés au SMIC,

est rédigé, un employeur ne pourrait jamais supprimer une prime, ce qui serait un non-sens. Le présent amendement vise donc à laisser la substitution jouer, dès lors que l'élément de salaire est supprimé avant l'attribution de la prime de partage.

Or, nous le savons bien, la hausse des prix frappe davantage nos concitoyens défavorisés et donc les bas salaires. C'est la raison pour laquelle nous proposons de prioriser le versement de la prime de partage de la valeur aux salariés dont les revenus sont les plus modestes, davantage exposés aux hausses de prix.

« il est expressément prévu que la prime de partage de la valeur ne puisse se substituer à aucun des éléments de rémunération, [ ...] ces dispositions semblent toutefois davantage relever d'une déclaration d'intention dépourvue d'une réelle portée normative. Il serait par ailleurs impossible d'aller vérifier, à l'occasion de chacun des versements, que la prime respecte bien cette condition de non-substitution ». C'est en

qui a permis de verser de manière agrégée 51 milliards d'euros de dividendes. Ces entreprises ont-elles réellement besoin d'être exonérées de cotisations sociales et fiscales pour verser des primes ? Quand allez-vous cibler et conditionner les aides, vous qui conditionnez et contrôlez le moindre euro de prestations sociales Les politiques d'exonération contribuent à normaliser les stratégies d'évitement fiscal et la tendance à ne pas prendre sa part dans la solidarité nationale.

d'une nouvelle décision unilatérale de l'employeur, tout en respectant la limite globale du plafond d'exonération. Cette possibilité n'étant pas prévue par les textes précédents, un tel choix était dépourvu de sécurité juridique. Le présent amendement a pour objet de donner une base légale à cette situation et de permettre aux entreprises qui en ont les moyens et la volonté de compléter leur prime de pouvoir d'achat au cours de l'année civile par une nouvelle décision unilatérale de l'employeur ou un nouvel accord d'entreprise dans la limite globale du plafond applicable et dans le respect des modalités initiales d'attribution. Ainsi, le caractère d'unicité de la prime est préservé.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Par cet amendement, nous demandons que les entreprises qui ont distribué des dividendes versent obligatoirement une prime de partage de la valeur aux salariés. Dès lors qu'une entreprise réalise des bénéfices, la logique de l'économie libérale voudrait qu'elle partage les profits avec ses salariés en premier lieu, avant de distribuer des dividendes aux actionnaires.

obligatoire le versement de la prime de partage de la valeur pour les entreprises qui ont versé des dividendes. Quel

Pour autant, leur résultat net agrégé a chuté de plus de 55 %. Ce rapport montre ainsi que ces entreprises se sont servi des aides publiques versées par l'État à faire face à la crise sanitaire pour rémunérer leurs actionnaires, tout en supprimant des emplois. Ces aides publiques- chômage partiel, prêts garantis par l'État, reports de cotisations sociales, plan de relance, plan d'urgence -ont été accordées sans aucune conditionnalité ou contrepartie sociale, fiscale ou environnementale et il est scandaleux que cet argent soit utilisé pour augmenter les profits d'une minorité. Le ministre Bruno Le Maire avait demandé à ces

qui en bénéficient prennent leur juste part de responsabilité face à l'urgence climatique, sociale et sanitaire. Afin de respecter nos engagements climatiques, les sociétés françaises doivent accélérer leur transformation dans le but d'être plus résilientes vis-à-vis des risques environnementaux. Cet amendement tend donc à favoriser leur transition rapide vers une économie bas-carbone. Elles doivent également prendre et respecter des engagements en matière de maintien de l'emploi et d'égalité entre les femmes et les hommes.

Le présent amendement prévoit qu'en cas de redressement le cotisant puisse s'exprimer physiquement devant la commission de recours amiable, s'il en émet le souhait.

Nous savons, parce que cela a été étudié depuis plusieurs années, que tout dispositif neutre en termes d'impact sur les femmes et les hommes est en réalité un dispositif qui, le plus souvent, accroît les inégalités de départ,

le voeu que le Gouvernement prenne plus au sérieux la question de la lutte contre les inégalités de genre et se dote des moyens d'améliorer sa politique

par les exploitants de remontées mécaniques à leurs employés pour les besoins du service sont considérées comme des avantages en nature, à hauteur de deux septièmes du prix du forfait de ski, et ce, alors même que l'utilisation de la carte durant les congés des employés n'est pas autorisée. À ce titre, ces cartes sont taxées par l'Urssaf, ce qui est illogique, puisqu'aucun avantage n'est consenti, les grilles tarifaires prévoyant déjà l'accès gratuit pour les jours de ski au-delà de vingt-cinq jours dans le forfait saison.

afin d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés et stopper des dépenses superflues et injustes pour ces derniers comme pour les exploitants de remontées mécaniques, cet amendement tend à supprimer la taxation réalisée par l'Urssaf des cartes de libre circulation utilisées par les salariés des domaines skiables.

l'amendement n° 124. Face à l'inflation, l'urgence sociale requiert des mesures fortes de revalorisation des salaires afin de permettre le maintien pérenne du pouvoir d'achat. Cela passe notamment par des accords de branche et d'entreprise dynamiques, prévoyant des augmentations de salaire, ainsi que par l'augmentation du SMIC.

l'amélioration des conditions de travail et/ou la revalorisation des salaires dans certains métiers ». En conséquence, le retour de l'attractivité de beaucoup de métiers et de branches passe par des rémunérations dignes et de meilleures conditions de travail,

c'est-à-dire les plus grandes d'entre elles -au titre des heures supplémentaires, poursuivant et accélérant la fuite en avant dans la réduction du salaire socialisé générateur de droits. Or ce nouveau dispositif d'exonération ne permet en rien d'aider les salariés ; il les contraint à toujours travailler plus pour espérer

à vous remercier

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

l'amendement n° 113 rectifié . Cet amendement de ma collègue Sylviane Noël a pour objet de redonner du pouvoir d'achat aux salariés, ce qui est bien l'enjeu du texte que nous examinons. Il vise à réduire le coût des heures supplémentaires et complémentaires pour les employeurs sans minorer la rémunération des salariés, puisque ces derniers continueraient de percevoir la majoration afférente aux heures supplémentaires. En revanche, les cotisations patronales de sécurité sociale seraient calculées sur la seule rémunération de base,

près d'1 milliard d'euros de pertes de recettes pour la sécurité sociale ! Même si l'État s'engageait à compenser cette perte de recettes pour la sécurité sociale, vous savez bien que c'est autant d'argent en moins pour les services publics. Le Gouvernement a trouvé une majorité pour le soutenir dans le « travailler plus pour gagner plus », mais votre proposition, c'est aussi moins d'emplois, moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins de services publics. Pour toutes ces raisons, nous demandons par cet amendement le maintien

Le scrutin est clos.

Mme Chantal Deseyne. Cet amendement vise à permettre le cumul de l'exonération partielle de cotisations sociales des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité en fonction des revenus des chefs d'exploitation. La modification proposée est nécessaire afin de permettre aux jeunes agriculteurs de bénéficier de la mesure prévue par le Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat des travailleurs indépendants.

Le code rural et de la pêche maritime permet à tous les chefs d'exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d'une modulation agricoles (Amexa). En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture et l'installation des jeunes, l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d'exploitation.

qui leur est réservée sont redevables, à revenu égal, de davantage de cotisations sociales que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la troisième année après l'installation, compte tenu du caractère dégressif de l'exonération partielle sur cinq ans. Cette anomalie doit être corrigée. Le présent projet de loi crée une mesure en faveur du pouvoir d'achat des travailleurs indépendants et renforce ainsi la modulation du taux d'Amexa.

dont le revenu est équivalent au SMIC. Si les travailleurs indépendants ont perdu durant la crise sanitaire en moyenne 10 % de revenus, le soutien du Gouvernement ne peut toujours se résumer à des exonérations ou des baisses de cotisations sociales. Nous voyons bien le piège, depuis la suppression d'une partie des cotisations sociales des employeurs au travers du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, de cette stratégie qui consiste à tirer vers le bas le montant des cotisations sociales.

Enfin, cette baisse de cotisations pour les travailleurs indépendants pose une sérieuse question d'équité depuis l'intégration des indépendants au régime général de sécurité sociale, ces derniers bénéficiant des mêmes prestations sociales, alors que leurs taux de cotisation sont largement inférieurs. S'il faut améliorer la situation de ces travailleurs, cela

En tout état de cause, ce sont des sommes considérables qui méritent débat. Le Gouvernement est ouvert à l'idée de rendre contributives des cotisations acquittées dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Cela nécessite de travailler sur la question des retraites et ce n'est pas la même

plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collective. L'article 3 prévoit d'assouplir les conditions de mise en oeuvre d'un dispositif d'intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés et d'autoriser leur adoption par décision unilatérale de l'employeur, lorsque les délégués syndicaux ou les instances représentatives du personnel sont inexistants, ou bien en cas d'échec des négociations portant sur la mise en place d'un accord d'intéressement. Autrement dit, si dans une entreprise les représentants du personnel refusent l'instauration de l'intéressement pour privilégier une augmentation des salaires, l'employeur pourra s'asseoir sur le refus des organisations syndicales. Nous refusons pour notre part ce passage en force des employeurs par décision unilatérale. Attachés aux principes qui ont présidé à l'instauration de la sécurité sociale dans notre pays, nous considérons que le véritable partage de la valeur dans les entreprises, ce sont les cotisations sociales. Les salariés et les employeurs financent ensemble une caisse commune, la sécu, dont les prestations sociales sont la part socialisée du salaire. Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à l'article 3. La parole

d'un accord d'intéressement constitue une véritable négation du dialogue social, de l'implication des salariés dans la vie de l'entreprise et du rôle des organisations syndicales. Voilà pourquoi nous entendons supprimer cet article.

pour l'employeur de décider, seul, en cas de désaccord ou de carence, le mode de calcul et les règles de répartition entre les salariés d'un dispositif d'intéressement

Ce nouveau contournement du coeur de la compétence et de la légitimité des organisations syndicales est unanimement condamné par les organisations de salariés et contredit le discours sur un changement de méthode quant au respect des corps intermédiaires. social et économique (CSE) est obligatoire dans les entreprises de plus de onze salariés, c'est précisément parce que le dialogue social au sein des entreprises est crucial. Rappelons que le partage de la valeur ajoutée brute s'effectue d'abord et avant tout par la négociation annuelle obligatoire, la fameuse NAO, et que les accords collectifs d'intéressement ne peuvent s'y substituer. Les organisations syndicales sont garantes de cette non-substitution, ce qui justifie amplement le refus d'une décision unilatérale de l'employeur. À l'opposé de l'article 3 qui exonère l'employeur de sa responsabilité dans l'obtention d'un accord avec les syndicats, il aurait été plus conforme à l'esprit du dispositif d'encourager les entreprises à lever les freins à la désignation de représentants du personnel ou à la création d'instances représentatives, et à respecter sans la contourner la compétence exclusive des syndicats. Par le présent amendement, nous voulons rappeler que la mise en place d'un dispositif d'intéressement suppose des négociations préalables et conclusives avec un délégué syndical ou des organisations syndicales ou au sein du comité social et

l'administration met chaque année à la disposition de l'entreprise un formulaire de type Cerfa, préalablement rempli avec toutes les informations dont elle dispose déjà sur le compte de l'entreprise. L'entreprise n'aurait plus qu'à compléter ou amender ces informations pour instaurer un intéressement. En outre, cela permettrait aux entreprises qui n'ont pas encore connaissance de la possibilité dont elles disposent d'en être informées par l'administration.

Cohen. Cet amendement vise à soumettre à des cotisations maladie les sommes versées au titre de l'intéressement. Les exonérations de cotisations qui sont liées à l'intéressement coûtent déjà 1,7 milliard d'euros par an à elles seules. C'est un dispositif qui, selon nous, bloque l'augmentation des salaires et assèche les recettes de la sécurité sociale, même si les pertes sont compensées. Ces coûts viendront demain justifier le transfert de certaines missions de la sécu aux assurances privées. Pour mémoire, les soins hospitaliers représentent pratiquement 50 % des dépenses du système de santé et, parmi l'ensemble des soins hospitaliers, près de 90 % sont financés par la sécurité sociale. L'assurance maladie étant le principal payeur de l'hôpital,

Un couple s'est présenté au centre hospitalier des Sables-d'Olonne, en Vendée, avec un bébé en détresse respiratoire. Ils n'ont pas pu être pris en charge aux urgences faute de médecins et ont dû se rendre dans un autre hôpital, situé à quarante kilomètres. Cette forme de refus de soins est d'une extrême gravité. Poursuivre les exonérations de cotisations maladie, c'est prendre le risque que ce genre de situation se multiplie jusqu'à devenir la norme en moins de temps qu'il ne faut pour réaliser une mission flash À l'heure où les urgences hospitalières sont contraintes de fermer leurs portes le soir et le week-end en raison du manque de personnel, car celui-ci ne supporte plus les conditions de travail dégradées dues en premier lieu au manque de moyens financiers,

parole est à Mme Corinne Féret. Par cet amendement, nous proposons de supprimer l'alinéa 4. En effet, il y a une contradiction intrinsèque dans la mise en oeuvre d'un régime d'intéressement sans accord ou ou consultation des organisations syndicales, puisqu'il s'agit d'impliquer et d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise. On créerait donc un dispositif d'implication des salariés sans les associer à la décision de mise en oeuvre dudit dispositif. Permettre à cette condition intrinsèque de perdurer jusqu'à cinq ans est excessif. Cinq ans, c'est long dans la vie d'une entreprise. Il convient que le dialogue social puisse retrouver sa place dans un délai plus court. Par ailleurs, la durée initiale d'homologation des dispositifs d'intéressement unilatéraux a été fixée à trois ans, au motif que les TPE-PME ne pouvaient pas forcément définir sur une longue période une formule de calcul sur la base d'indicateurs pertinents, par manque de prévisibilité à moyenne échéance de leurs résultats. Ce motif est toujours valable.

que leur secteur soit pourvu d'un accord de branche ou pas. L'intéressement est un dispositif facultatif. Les branches l'ayant mis en place par accord collectif proposent aux entreprises un dispositif clé en main, qu'elles sont libres d'utiliser ou pas. Ces dernières peuvent toutefois souhaiter mettre en place l'intéressement en choisissant des dispositions différentes de celles définies par la branche. Il est donc regrettable qu'une entreprise de moins de cinquante salariés appartenant à un secteur pourvu d'un accord de branche ne puisse pas décision unilatérale de l'employeur (DUE). Lorsqu'il existe un accord de branche agréé, les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter par DUE pour l'application directe du dispositif de branche. faculté n'est toutefois laissée que dans la mesure où l'entreprise reste dans le cadre des options préfixées par les branches. Une entreprise de moins de cinquante salariés qui ne trouverait pas dans l'accord de sa branche la formule d'intéressement convenant à sa situation ne pourrait donc donc pas mettre en place un intéressement par DUE, alors que cette possibilité serait ouverte à l'entreprise dont la branche n'a pas négocié. Quel est l'avis de la commission

L'article 3 prévoit que, si l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale de l'employeur pour une durée comprise entre un an et cinq ans. Afin de Afin de favoriser le dialogue social dans l'entreprise, il serait préférable que la durée maximale ne soit pas aussi longue. Nous proposons donc de la raccourcir à trois ans. Cette durée nous semble suffisante pour que l'entreprise et les représentants des salariés discutent et conviennent d'un nouvel accord d'intéressement.

de la suppression de l'article 3. Ils ont pour objet de reconnaître toute sa place au dialogue social dans l'entreprise. Celui-ci vise à compléter l'alinéa 8 pour limiter la faculté d'imposer un dispositif d'intéressement aux seules entreprises qui respectent leurs obligations en matière de représentation du personnel. Il s'agit d'éviter que des entreprises dans lesquelles l'absence de CSE serait de la responsabilité de l'employeur ne puissent utiliser la procédure dérogatoire d'homologation d'un accord d'intéressement unilatéral. Nous voulons donc limiter cette procédure aux entreprises vertueuses.

cet amendement vise à supprimer la possibilité pour l'employeur d'imposer par la force la mise en place de l'intéressement, y compris en cas d'échec des négociations. Cette brèche ouverte dans l'équilibre fragile des rapports entre l'employeur et les représentants du personnel nous semble particulièrement dangereuse.

tenu de la place structurelle que tendent à prendre les rémunérations hors salaire dans la rémunération globale, il ne nous semble pas acceptable que l'employeur puisse passer outre à la volonté des salariés. Quel

Cet amendement vise à étendre la date limite de conclusion de l'accord d'intéressement au dernier jour du troisième trimestre, contre le dernier jour du deuxième trimestre actuellement. Grâce à cet assouplissement, les entreprises auraient davantage de temps pour négocier leurs accords. Par ailleurs, l'intéressement gagnerait en efficacité, car le délai entre le moment où l'intéressement est mis en place et celui où il produit des effets serait raccourci.

L'objectif est d'encourager les entreprises à mettre en place de tels accords. Le montant de cet intéressement d'amorçage est limité à 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Il sera pris en compte dans les plafonds applicables aux primes d'intéressement et sera soumis au même régime L'octroi de cet intéressement d'amorçage sera possible pour toute conclusion d'un nouvel accord d'intéressement, à condition qu'aucun accord d'intéressement n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet du nouvel accord.

commission

pour les salariés et les entreprises. Ils permettent de partager la valeur créée par l'entreprise, lorsque certains objectifs sont atteints, s'agissant de l'intéressement, ou en fonction du résultat d'une formule de calcul, de la participation. Les entreprises peuvent également abonder volontairement les plans d'épargne salariale de leurs salariés. Ces dispositifs sont encouragés par des régimes fiscaux et sociaux spécifiques. Ils sont favorables au pouvoir d'achat des salariés.

à leur diffusion. Alors que le partage de la valeur et des gains de pouvoir d'achat doit être intensifié et stimulé, il est nécessaire d'harmoniser les taux de forfait social et de simplifier leur fonctionnement. Pour encourager la mise en place de ces mécanismes de partage de la valeur au bénéfice des salariés, cet amendement vise à harmoniser les régimes, en exonérant exonérant de forfait social l'ensemble de ces dispositifs. Cette mesure permettra, en outre, d'exonérer de forfait social la prime de partage de la valeur instituée par l'article 1 de ce projet de loi. En effet, à la différence de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA), à laquelle elle succède, cette prime est soumise au même forfait social que l'intéressement.

Le principe consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise ou représentant une quote-part de ses bénéfices. Les sommes attribuées peuvent, selon le choix du salarié, lui être versées directement ou être déposées sur un plan d'épargne salariale. Ces dispositifs sont encouragés par des régimes fiscaux et sociaux spécifiques et sont favorables au pouvoir d'achat des salariés. La multiplication des taux, selon le dispositif concerné et selon la taille de l'entreprise, engendre une situation complexe, dépourvue de lisibilité et d'harmonisation, créant de surcroît des effets de seuil. Cet amendement vise donc à harmoniser l'ensemble des régimes, en exonérant de forfait social ces dispositifs dès lors que l'entreprise compte moins de 250 salariés.

Cette exonération permet d'inciter les salariés à diriger leur épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises, d'accroître l'actionnariat salarié- un facteur de motivation et de fidélisation des salariés -et ainsi de favoriser le partage de la valeur dans l'entreprise. La présente proposition a pour objet de proroger l'exonération temporaire de forfait social

qui complètent les versements des salariés pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise ou d'une entreprise du groupe. Cette exonération permet d'inciter les salariés à diriger leur épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises, d'accroître l'actionnariat salarié- salarié- un facteur de motivation et de fidélisation des salariés -et ainsi de favoriser le partage de la valeur dans l'entreprise. La présente proposition a pour objet de proroger l'exonération temporaire de forfait social prévue par la loi de finances initiale pour 2021 jusqu'au 31 décembre 2024.

produit. Il est disponible depuis le 1 octobre 2019 et remplace les autres plans d'épargne retraite. Ce produit d'épargne est composé de trois types de versements : les versements individuels, l'épargne salariale et les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur. Lors du départ à la retraite, les versements peuvent être récupérés, soit en capital, soit en rente viagère, à l'exception des versements obligatoires qui ne peuvent être délivrés que sous forme de rente viagère. Cet amendement tend à laisser au titulaire de l'épargne la possibilité de choisir son mode de liquidation,

et des congés payés au-delà de la cinquième semaine de congés payés est aujourd'hui possible pour les entreprises couvertes par un accord collectif dans le cadre d'un compte épargne-temps L'article 6 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes, ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avait permis une monétisation simplifiée des jours de repos conventionnels et d'une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, et ce de manière exceptionnelle jusqu'au 30 juin 2021. Il serait souhaitable que cette monétisation simplifiée soit pérennisée pour les jours

qui gagnent jusqu'à deux fois le SMIC peuvent bénéficier d'une aide carburant de 40 euros par mois, financée à 50 % par l'employeur volontaire et à 50 % par le conseil régional. Ce dernier signe une convention avec l'entreprise

ou d'alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements domicile-travail. Ce dispositif est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite de 310 euros par an. Les auteurs de l'amendement proposent d'augmenter ce plafond à 500 euros par an,

donc un signal fort et un accompagnement financier intéressant pour les salariés, dont la baisse inquiétante du pouvoir d'achat doit être limitée autant que possible. Ce dispositif est par ailleurs un bon moyen de sortir de l'autosolisme. Près de 75 % des employés qui vivent à moins de 5 kilomètres de leur travail se déplacent en voiture. Notre part modale du vélo reste scotchée à 4 quand l'Allemagne atteint 12 %. Il est donc temps d'actionner ce levier déterminant, dont les avantages sont nombreux : un moyen de transport économique, peu polluant, idéal pour décongestionner les villes, excellent pour la santé, et même pour la productivité- des employeurs ayant mis le FMD en place en attestent. Ce forfait a fait ses preuves. Il s'agit à présent de le généraliser afin qu'il produise de façon

Il souligne que les bons sociaux sont des instruments puissants pour augmenter les recettes fiscales de l'État, stimuler la création d'emplois et augmenter le pouvoir d'achat des salariés, tout en développant l'économie locale. Le titre-restaurant, par exemple, est un dispositif social performant qui rapporte plus qu'il ne coûte à l'État. S'appuyant sur ce rapport, il est proposé de mettre en place un forfait télétravail qui permettrait à l'employeur de prendre en charge tout ou partie des frais générés par le télétravail, selon ce même principe de titres fléchés, qui répond également à un besoin lié au développement durable. Les bénéficiaires seraient les salariés des entreprises du secteur privé et les agents du secteur public ou des groupements d'intérêt public. Lorsque l'entreprise décide d'accorder cette aide financière, son montant et ses modalités d'attribution seraient déterminés par accord d'entreprise, par accord interentreprises, ou à défaut par accord de branche ou au niveau des comités sociaux et économiques. La mise en oeuvre du forfait télétravail par décision unilatérale de l'employeur serait subordonnée à la consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe. Quel est l'avis de la commission ? Je remercie

du Gouvernement ? Il est défavorable. Les frais engagés lors du télétravail relèvent du régime juridique des frais professionnels et la prise en charge par l'employeur des coûts liés à l'exercice des fonctions est une obligation générale issue de la jurisprudence, dont il ne peut s'exonérer.

Le titre-restaurant est connu et utilisé par des millions de travailleurs. Il permet notamment aux salariés à faibles revenus de diviser par deux le coût de leur pause déjeuner. Il est également fiscalement avantageux pour les entreprises, générateur de chiffre d'affaires pour les commerçants

Pour être exonérée des cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre ; par ailleurs, elle ne doit pas excéder un certain montant. à 7,50 euros permettrait donc indirectement d'augmenter le ticket journalier à environ 15 euros. Depuis le 1 janvier 2020, la limite d'exonération n'est plus la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu, mais la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1 octobre de l'avant-dernière année et le 1 octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant. Cette valeur maximum s'élève à 5,69 euros pour 2022. Il suffirait d'augmenter le plafond maximal des sommes versées chaque jour travaillé par les entreprises à leurs salariés, et par conséquent la participation patronale, pour contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat et la qualité de l'alimentation.

voeux porterait, d'une part, sur la possibilité d'élargir les bénéficiaires des titres-restaurant et, d'autre part, sur la possibilité de mettre en place de nouveaux titres fléchés répondant à l'objectif que je viens de rappeler. Quel est

L'enjeu est réel : la non-répercussion de l'évolution du SMIC dans l'échelle des salaires contribue à compresser les écarts entre les différents niveaux de la grille et à élargir les effectifs proches des minima de branche, neutralisant

très raisonnable -suivant la seconde revalorisation du SMIC. Les deux

de restructurer une branche. La difficulté structurelle pour une branche de conclure un accord garantissant que ses minima soient au niveau du SMIC devenait ainsi un indice de la faiblesse de la vie conventionnelle d'une branche.

d'un projet de fusion et de restructuration de la branche. Cette dernière aurait alors deux solutions : soit réagir immédiatement en ouvrant des négociations pour se mettre en accord avec la loi, soit se soumettre à la restructuration ainsi prévue.

sont encore dans cette situation, ce qui signifie que 55 ont fait le travail de négociation depuis le 1 mai jusqu'à aujourd'hui. La nouvelle revalorisation du SMIC le 1 août entraînera une situation assez identique à celle du 1 mai, avec de nouveau des ouvertures de discussion. l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise à réduire de 90 à 45 jours le délai au cours duquel les branches doivent ouvrir des négociations, si un minimum passe en dessous du SMIC, ce qui dynamiserait encore plus le dialogue social. Je ne dis pas que l'outil est parfait,

pour limiter le mécontentement des salariés, voire leur départ, les gouvernements ont usé d'un mélange d'augmentations individuelles et de primes de vie chère. Ils ont rejeté l'idée d'une indexation, en maintenant la décentralisation de la fixation des salaires. En 1952, l'échelle mobile des salaires fut adoptée, sous la présidence de Vincent Auriol, avant d'être malheureusement supprimée en 1982. Maintenir automatiquement chaque année le pouvoir d'achat des travailleurs salariés est une mesure de justice élémentaire. C'est un outil parmi d'autres, qui soutiendrait le dynamisme de notre économie. Des mécanismes d'indexation existent pour certaines prestations familiales, pour les retraites ou encore pour le SMIC. Pourquoi pas pour tous les salariés ? Tel était d'ailleurs le sens d'une proposition de loi déposée par nos collègues de l'Assemblée Voilà plusieurs semaines que l'inflation, autrement dit la hausse globale des prix, a relancé le débat sur l'urgence d'augmenter les salaires. Pour neutraliser la diminution mécanique du pouvoir d'achat des salariés, il est nécessaire de la compenser. Le rétablissement Le rétablissement d'une échelle mobile des salaires permettrait de garantir une augmentation automatique de ceux-ci en fonction de l'augmentation des prix, afin que soit durablement préservé le pouvoir d'achat des salariés. L'amendement

Madame le rapporteur,

en situation de pauvreté que les hommes : entre 18 ans et 49 ans, les écarts de taux de pauvreté sont compris entre 1,9 point et 3,8 points. Ces différences s'expliquent principalement par un nombre plus important de mères isolées. Les familles monoparentales présentent des taux de pauvreté très élevés-

Les différentes rustines gonflées à l'argent public ne suffisent plus à résorber la baisse du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Plutôt que de parler de primes, la proposition du groupe SER vise à parler de salaires. de salaires. À cet effet, nous vous proposons, monsieur le ministre, de convoquer un Grenelle des salaires. La nécessité d'une grande concertation nationale sur les salaires, secteur par secteur, type d'activité par type d'activité, type de contrat par type de contrat, est non plus une option, mais une obligation.

et le capital. Le contexte inflationniste appelle des mesures d'urgence. C'est précisément cette urgence qui préside à la demande de la tenue d'un Grenelle des salaires dès la promulgation de la loi

amendement vise à rendre obligatoire l'ouverture des négociations pour l'ensemble des minima conventionnels de branche, dont ceux des cadres, lorsque le SMIC fait l'objet d'une seconde revalorisation dans la même année. année. Pour se mettre en conformité avec le niveau du SMIC, de nombreuses branches se contentent en effet de procéder à des revalorisations qui ciblent uniquement le bas de la grille salariale. Quelques-unes suppriment ainsi uniquement les coefficients immergés. Par conséquent, Par conséquent, la non-répercussion de l'évolution du SMIC sur l'ensemble de l'échelle des salaires participe à compresser les écarts entre les différents niveaux de salaires, d'où un risque important de déclassement, notamment pour les cadres. Afin d'inciter les branches à conclure des accords salariaux pour l'ensemble des minima conventionnels de branche, cet amendement vise à ajouter une conditionnalité aux allègements généraux de cotisations patronales. Il s'agirait, si je puis dire, d'une véritable menace. Il est ainsi proposé de suspendre le bénéfice des allègements généraux de cotisations patronales en cas d'absence de revalorisation des minima conventionnels de branche. Cette suspension interviendrait six mois après la date de la seconde revalorisation du SMIC, un délai raisonnable. Elle pourrait être levée à la date de signature de l'accord de revalorisation, avec un effet rétroactif des allègements de cotisation patronale sur la période de suspension. Cet amendement vise donc à freiner le phénomène de resserrement de l'éventail des

de branche. Dès lors que les minima seraient inférieurs au SMIC pendant plus de six mois, les entreprises ne pourraient plus bénéficier des exonérations de cotisations sociales applicables. Si les négociations de branches devaient déboucher dans ce délai, ce bénéfice serait

coefficient inférieur au SMIC en vigueur, après la revalorisation de celui-ci en mai dernier. Certes, ce découplage s'explique en partie par les hausses successives automatiques du SMIC. Pour autant, certaines branches se sont rapidement conformées à la hausse, notamment dans une optique d'amélioration de l'attractivité des métiers concernés. C'est notamment le cas de l'hôtellerie-restauration, qui a récemment augmenté sa grille de 16 % en moyenne, avec des minima au-dessus du SMIC. Par cet amendement, nous proposons d'accélérer les négociations en faveur du pouvoir d'achat des salariés, en retirant le bénéfice des réductions de cotisations sociales aux branches dont les minima restent en dessous du SMIC durant l'exercice social où ces revalorisations du SMIC ont eu lieu. Nous rendons efficace le mécanisme de sanctions inclus dans le présent projet de loi, afin d'accélérer le rattrapage du SMIC par les branches sans pénaliser les entreprises, tout en offrant une solution efficace à la protection du pouvoir d'achat, qui suppose une démarche d'augmentation des salaires. Le conditionnement des réductions de cotisations sociales à l'obligation d'afficher des minima de branche supérieurs au SMIC est un levier qui permettrait de stimuler efficacement les négociations de branche, dont l'importance est majeure,

Monsieur le ministre, 318 qui prévoit une conditionnalité des exonérations, il existe une difficulté de mise en oeuvre. Une telle disposition avait été adoptée en 2008, mais elle n'a jamais été appliquée dans la mesure où il suffirait qu'une branche ne procède pas à la négociation rendue obligatoire par la loi pour que les entreprises de la branche perdent le bénéfice de l'exonération. Cela signifierait qu'une entreprise pratiquant une politique salariale à un niveau supérieur aux minima conventionnels de sa branche serait sanctionnée du fait de la défaillance de la branche à laquelle elle appartient.

Initialement, les allègements de cotisations patronales visaient à favoriser l'embauche de salariés peu qualifiés. Malheureusement, ce dispositif semble parfois être dévoyé, ces allègements incitant certaines entreprises à ne pas augmenter les salaires. Aussi, nous proposons de mettre un terme au bénéfice de ces allègements, dès lors que les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté ont une rémunération égale au SMIC. Cette mesure participerait à l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires les plus modestes.

des effets néfastes pour les salariés. Elle joue en effet un rôle majeur dans le maintien et l'extension des bas salaires. Les entreprises étant incitées à ne pas augmenter les salaires, de très nombreux salariés se voient maintenus durant plusieurs années à des salaires avoisinant le SMIC.

Par cet amendement, nous souhaitons conditionner les aides publiques pour les grandes entreprises à la conclusion d'un accord avec les représentants des organisations syndicales. Nous proposons de favoriser la conclusion des accords de branche dans les six mois suivant le début des négociations. Afin que le sujet du salaire minimum par branche progresse de façon rapide et durable, il convient, sinon de contraindre, du moins d'inciter à mener à bien ces négociations dans un délai raisonnable, en faisant dépendre de leur réussite l'attribution des aides publiques aux entreprises. Par ailleurs, l'amendement tend à réduire de quatre ans à deux ans le délai obligatoire

fixés juste au-dessus du SMIC ne passent pas automatiquement en dessous, entretenant ainsi la spirale des bas salaires et le tassement des rémunérations.

des droits au salarié, le salaire net n'étant qu'une partie de la rémunération du travail. Éviter la part socialisée revient de fait à baisser la rémunération.

C'est aussi l'un des visages de la précarité. Or, comme l'inflation s'inscrit très certainement dans la durée, ses effets sur le pouvoir d'achat ne seront durablement amoindris que par une réelle augmentation de la rémunération fixe, garante d'un renforcement de la résilience sur le temps long de l'ensemble des salaires, notamment

les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation de la révision des salaires prévue par ces conventions ou accords ». Du reste, il me semble qu'il n'appartient pas au ministre du travail d'ordonner aux partenaires sociaux de conclure un accord. L'avis de

un rapport au champ de réflexion étendu sur les rémunérations, les conditions de travail, le parcours professionnel, les qualifications, mais aussi la répartition de la richesse. Elle serait composée non pas seulement de macroéconomistes, et de représentants des partenaires sociaux. L'avantage d'une telle composition est de réunir tous les acteurs, en articulant compétences techniques et politiques. Cette commission pourra s'appuyer sur les services de l'administration et les institutions productrices de données utiles à ses travaux.

des représentants des organisations syndicales et des membres des organisations et associations travaillant dans le champ de l'insertion et du travail. Cela permettrait d'avoir une instance plus représentative de la diversité des expertises nécessaires à une étude plus complète et plus objective. Aujourd'hui, ce groupe est exclusivement constitué d'économistes qui appartiennent tous à la même école de pensée, il rend donc des rapports aboutissant à la même conclusion : une sous-indexation du SMIC. Cette modification de la composition du groupe d'experts permettrait d'aboutir à une augmentation du pouvoir d'achat des salariés au SMIC.